publication de la loi. Tel qu'il est issu de l'examen en commission des affaires économiques, l'alinéa 11 exclut du champ de cette interdiction les oiseaux de voleries itinérantes.

Buis. Cet amendement vise à supprimer les modalités de rédaction du décret fixant une liste d'animaux domestiques dont la détention est interdite dans les établissements itinérants. Dans la pratique, les critères régissant cette interdiction se révèlent complexes et cumulatifs. Dès lors, cette liste devient difficile à élaborer, ce qui pourrait avoir pour conséquences de rendre la disposition inopérante et d'augmenter les risques de fragilités juridiques en cas de contentieux. De plus, l'article réécrit par la commission crée une instance chargée de rendre un avis sur le projet de décret fixant la liste des espèces animales non domestiques interdites de présentation au public en établissement itinérant. Or deux instances consultatives compétentes peuvent déjà rendre un tel avis : le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive

le Conseil constitutionnel s'assure que les critères justifiant la restriction d'une liberté sont suffisamment détaillés. En les supprimant, on fragiliserait le présent texte. J'ajoute que je suis prête à réfléchir à la fusion du comité proposé avec la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

à revenir sur l'obligation faite à tous les spectacles présentant des animaux non domestiques de revêtir une dimension pédagogique, et seulement celle-ci. Il s'agit là d'un point essentiel, de nature à faire véritablement évoluer le contenu des présentations tout en créant un lien plus fort entre l'homme et l'animal.

de vétérinaires spécialistes de la faune sauvage captive, plus exactement des animaux non domestiques captifs. Or ces personnes sont en conflit d'intérêts absolu : c'est leur métier, c'est leur gagne-pain ! Comment faire prévaloir l'avis

Vous préférez laisser la décision à des vétérinaires qui ne sont pas spécialistes de la faune sauvage captive ; pour ma part, je considère qu'ils peuvent parler mieux que quiconque des sujets qui les concernent.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Dans les océans, il est habituel de les voir parcourir jusqu'à 100 kilomètres par jour et plonger à des profondeurs atteignant 200 mètres. Ils sont presque toujours en mouvement. Même lorsqu'ils se reposent, ils passent moins de 20 % de leur temps à la surface de l'eau. Dans les delphinariums, les dauphins se retrouvent brutalement enfermés entre quatre murs de béton, dans une eau traitée chimiquement, souvent au moyen de chlore- il est donc impossible d'introduire des poissons vivants ou des algues dans leurs bassins. La privation de liberté rend les dauphins malades, stressés, dépressifs. L'espérance de vie des dauphins sauvages est, en moyenne, de 45 ans pour les mâles et de 55 ans pour les femelles. En revanche, leur espérance de vie en captivité n'est que de 20 ans,

En liberté, leur régime alimentaire est très varié. En captivité, le dauphin est nourri de poissons morts massivement enrichis de vitamines et d'antibiotiques. Quelles que soient les conditions d'accueil que l'on réserve aux cétacés, quels que soient les efforts déployés pour élargir encore la taille des bassins, leur enfermement n'en reste pas moins, toujours et dans tous les cas, contre-nature. À travers cet amendement, il nous paraît également primordial de rétablir l'interdiction de leur reproduction,

nous estimons qu'il faut aller plus loin que les seuls garde-fous adoptés en commission. Ainsi, cet amendement tend à reprendre les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale concernant les mesures d'interdiction de détention des cétacés en captivité, les certificats de capacité et autorisations d'ouverture correspondantes et les entrées en vigueur, en apportant quelques modifications pour gagner en clarté.

l'on peut interdire les spectacles en tant que tels, il ne faut pas interdire leurs activités. Nous devons donc autoriser des présentations à but pédagogique, qui utilisent les comportements spontanés des cétacés. C'est une façon raisonnable, équilibrée, mais ferme de traiter cette question afin que nous puissions enfin en voir la fin.

d'interdire la détention. Il faut effectivement prévoir des refuges de nature marine, où ces animaux puissent retrouver un milieu proche de leur milieu naturel.

la plus équilibrée : à savoir la possibilité d'interdire par décret la détention et l'acquisition de cétacés, mais au regard de critères stricts et suivant l'avis d'un conseil spécialisé. C'est le rôle du Sénat de définir précisément les critères justifiant une telle interdiction et de fonder toujours ses décisions sur des expertises scientifiques, pour le bien-être des animaux, au cas par cas, plutôt que de formuler une interdiction générale de principe.

et ainsi de rendre plus difficile leur prise en charge à l'issue de ce dispositif. Les orques, par ailleurs, ne se reproduisent pas en captivité. Les delphinariums maîtrisent en revanche déjà la reproduction des dauphins.

soustraire la France de ce programme de recherche, qui tend à étudier la perception par les dauphins des ondes magnétiques, leur communication, ou encore d'autres éléments susceptibles de nous aider à mieux les protéger me paraîtrait être une erreur.

voix l'amendement n° 176. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

effet, le décret d'interdiction des cétacés et celui établissant la liste des espèces d'animaux non domestiques interdites dans les établissements itinérants devront prendre en compte l'existence de capacités d'accueil des animaux dans des conditions qui ne peuvent pas être moins favorables que dans les établissements de

De même qu'il existe un cadre légal pour les fourrières, les refuges et les centres de soins pour les animaux domestiques et les animaux sauvages indigènes, il est important d'en définir un pour les structures d'accueil d'animaux non domestiques non indigènes. Quel est l'avis de la commission ? Il me Il me semble essentiel de distinguer les trois modalités d'accueil des animaux, à savoir les refuges et les sanctuaires, appellations de plus en plus utilisées, parfois sans fondement, et les centres de soins pour faune sauvage déjà bien encadrés

doit être étudiée dans le cadre d'un travail réglementaire conduit avec les professionnels concernés. Une définition établie en concertation avec tous les acteurs doit s'imposer avant toute inscription dans la loi. Tel est le sens de cet amendement. L'amendement n° 73 rectifié,

les centres de soins de la faune sauvage sont déjà définis dans la réglementation, par l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage. Comme je l'ai dit pour les refuges et les sanctuaires, une définition par voie réglementaire, en favorisant la souplesse,

Au regard des conditions de fonctionnement des lieux de divertissement que sont les discothèques ou les plateaux des émissions de télévision, la présentation d'animaux non domestiques n'est jamais compatible avec leurs impératifs biologiques. Il n'est donc pas utile de limiter l'interdiction à une liste d'espèces fixée par arrêté. Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer la référence à la « vocation pédagogique », car je ne suis pas certain que les discothèques puissent avoir des visées pédagogiques à l'encontre des espèces animales

ou dont l'accès est restreint, dont la vocation première est d'accueillir du public, même dans le cadre d'événements privés, en vue d'un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse, sans vocation pédagogique ». Le présent amendement vise à supprimer le critère relatif à la vocation pédagogique, facilement contournable et superfétatoire.

Les ours et les loups ont des impératifs biologiques qui ne sont pas compatibles avec la détention et avec des spectacles nécessitant un dressage. Celui-ci provoque des mouvements stéréotypés, qui traduisent une maltraitance de ces animaux.

et qu'ils sont transportés au gré des évènements au cours desquels ils sont présentés. Il me semble donc que la rédaction proposée permet bien de caractériser ces deux activités, qui sont, en réalité, assez différentes.

15, dans sa rédaction actuelle, interdit uniquement l'élevage de visons et les élevages d'animaux d'espèces non domestiques. Cette rédaction restrictive n'empêcherait donc nullement la production de fourrure à partir, par exemple, Cet amendement vise donc à élargir l'interdiction de l'élevage à l'ensemble des animaux destinés exclusivement à la production de fourrure. Cette disposition n'aurait pas d'impact dans l'immédiat, dans la mesure où, à l'heure actuelle, seuls les visons sont élevés spécifiquement dans ce but, mais elle interdirait que, à l'avenir, quelqu'un se mette en tête de lancer un élevage de lapins ou de tout autre animal à fourrure. Cette rédaction ne faisant pas de distinction entre animaux domestiques et animaux non domestiques, elle a un caractère plus universel que la rédaction actuelle. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement tend

Sur le fond, si l'on se lance dans une série d'interdictions en visant les lapins consommés également pour leur chair, où sera la limite ? Qu'en sera-t-il des lapins consommés pour leur chair et qui découlent génétiquement du lapin angora ?

Pour ma part, je pense que le délai d'adaptation doit être suffisant. Une transition agricole prend du temps, des investissements doivent être réalisés. Je vous laisse vous mettre à la place des éleveurs : ils sont jugés, insultés, brimés et des associations pénètrent dans leur domicile la nuit.

études statistiques, qui montrent que l'apparition du variant, en Italie, au début de la pandémie, est géographiquement très liée à la présence de trois immenses élevages de visons dans la région contaminée en premier.

Cet amendement tend à prévoir un régime de sanctions en cas de méconnaissance des interdictions prévues dans le texte issu de l'examen du Sénat.

traitant de la fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. Ces sanctions s'élèveraient à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende. Cela permettrait de donner toute leur force coercitive aux dispositions que nous avons adoptées. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement

La maltraitance est insupportable ; il est de notre responsabilité de la combattre et nous le faisons. Par ailleurs, le lien humain avec les animaux est primordial pour lutter contre leur souffrance

proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Je rejoins ce qui vient d'être dit, la question de la maltraitance n'est pas exactement la même chose que le bien-être animal. Lorsque nous aurons mis

nommons les choses avec les bons mots. Nous proposons donc de rédiger ainsi l'intitulé du texte : « proposition de loi initiant les premières mesures contre la maltraitance animale » afin de préciser que les mesures adoptées dans le cadre de ce texte, aussi nécessaires soient-elles, ne constituent qu'une première étape.

explication de vote. Ce texte était nécessaire pour améliorer la condition animale, mais il n'est pas suffisant. Il est clair, par exemple, qu'un texte contre la maltraitance animale devrait inclure

La Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA) a actualisé en 2018 la Déclaration universelle des droits de l'animal de 1978 pour qu'elle puisse être adoptée par les législateurs dans des termes de droit positif juridiquement valides et effectivement applicables. Cette déclaration comporte huit articles, qui peuvent faire l'objet d'une proposition de résolution venant utilement compléter la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui.

certains de ses articles s'appliquent à tous les animaux. En outre, chaque article est rédigé comme un article de loi. Il ne s'agit pas d'un préambule théorique, mais d'une liste de principes parfaitement cohérente avec l'opinion très majoritaire des citoyens de notre pays.

vote. La protection des animaux n'est pas une préoccupation nouvelle, mais la demande sociétale est forte aujourd'hui et le sujet nécessite sans doute de moderniser notre cadre législatif. La proposition de loi que nous avons examinée vise un périmètre restreint, elle se concentre essentiellement sur la lutte contre la violence et la maltraitance exercées sur les animaux. Elle contenait, à l'issue de son examen à l'Assemblée nationale, des mesures positives. Mais elle proposait également des mesures qui n'étaient pas en phase avec la réalité des pratiques, voire totalement dogmatiques : certaines étaient inabouties ou déjà satisfaites par le droit existant, d'autres auraient fragilisé les acteurs de terrain, au détriment des animaux et, bien évidemment, de leur bien-être. C'est pourquoi le Sénat a privilégié une approche constructive, avec des solutions opérationnelles élaborées en lien avec les professionnels,

ses propositions, à lutter contre les abandons avec, par exemple, la mise en place d'un délai de réflexion de sept jours avant l'acquisition d'un animal, à maintenir les activités des animaleries pour ne pas favoriser le développement de réseaux de vente non contrôlés tout en encadrant leurs activités, faciliter et encadrer le recours aux familles d'accueil d'animaux abandonnés, à donner un véritable statut aux associations sans refuge, à renforcer le cadre de la vente des animaux sur internet, devenu la première animalerie, à refuser la compétence obligatoire du maire en matière de capture, d'identification et de stérilisation des chats errants sans moyens supplémentaires octroyés par l'État,

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la troisième session extraordinaire de 2020-2021.